visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels est parvenue à l'adoption d'un texte commun. J'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein des commissions mixtes paritaires chargées d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi organique et de la proposition relative aux lois de financement de la sécurité sociale ont été publiées.

À la demande du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, le Sénat a inscrit à l'ordre du jour ce débat sur les droits des personnes en situation de handicap. Il nous a semblé important et utile d'avoir, à six mois de l'élection présidentielle et des élections législatives, une discussion dans notre Haute Assemblée sur l'effectivité et le respect des droits des personnes en situation de handicap. Nous aurons, le 12 octobre prochain, l'occasion d'aborder une nouvelle fois la question de l'individualisation de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et de débattre avec le Gouvernement de la nature de cette allocation. L'AAH est-elle un revenu minimum de subsistance octroyé par l'État, calculé selon le foyer familial, ou une véritable prestation sociale de compensation du handicap individualisée, selon la situation propre du demandeur ? Pour notre part, la réponse est évidemment la seconde. Sans la déconjugalisation, que nous sommes nombreuses et nombreux ici à soutenir, il est impossible de sortir d'une situation de dépendance. En effet, notre société enferme en particulier les femmes en situation de handicap qui vivent en couple : 75 % d'entre elles se sentent dépendantes de leur conjoint. De surcroît, on estime que 34 % des femmes en situation de handicap en France ont subi des violences physiques ou sexuelles de la part d'un partenaire ou d'un ex-partenaire. Tout en abordant la question des aides financières, notre objectif est donc de mener une réflexion globale sur les personnes en situation de handicap, en partant de leurs droits et de leur mise en oeuvre effective au quotidien. En effet, la crise sanitaire a mis à rude épreuve notre système de protection sociale. Selon l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, elle a exacerbé les inégalités des publics vulnérables, tels que les personnes en situation de handicap. Avant toute chose, il faut rappeler qu'il y a, d'un côté, le handicap et, de l'autre, la personne en situation de handicap. Il ne faut pas les confondre. En France, une personne sur quatre souffre d'une incapacité, d'une limitation d'activité ou d'un handicap.

Le 14 septembre 2021, le Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies a rendu son rapport sur la mise en oeuvre, par la France, de la convention relative aux droits des personnes handicapées. Il a fortement critiqué le système actuel, qui prévoit des réponses isolées pour les personnes concernées et perpétue la méprise selon laquelle les personnes handicapées seraient objets de soins et non pas sujets de droit.

L'ONU estime que la France adopte un modèle médical et des approches paternalistes du handicap, qui nuisent à la bonne application des droits des personnes handicapées.

Notre société doit repenser son approche du handicap dans notre pays. Pourtant, la France avait fait un premier pas en ce sens lors de l'adoption de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Cette loi reconnaissait pour la première fois la responsabilité de l'environnement dans la production du handicap et traitait de la compensation, par le biais de prestations ou de services, en posant le principe de l'accessibilité à tout, pour toutes et tous. Malheureusement, depuis 2005, les gouvernements successifs ont été incapables de tenir les engagements inscrits dans la loi. Si des avancées ont pu avoir lieu, nous sommes encore très loin d'une société inclusive. Il suffit de constater l'absence de publication de certains décrets pour se convaincre que l'accessibilité à l'école, à l'emploi

de concevoir une société où les biens et services sont accessibles à toutes et à tous et où toutes les citoyennes et tous les citoyens peuvent faire valoir leurs capacités en exerçant leurs droits fondamentaux. Dans un rapport du mois d'août, la Défenseure des droits a, elle aussi, fait état d'un bilan contrasté s'agissant de l'effectivité des droits des personnes en situation de handicap. Ainsi, en 2020, le handicap est, pour la quatrième année consécutive, le premier motif de saisine de la Défenseure des droits en matière de discrimination, ce motif Pendant la crise de la covid-19, les personnes en situation de handicap et leurs proches ont subi, comme souvent dans leur quotidien, hélas ! l'absence d'aide, de soutien et de répit. Face à ces constats alarmants, construire une société inclusive et solidaire s'impose, c'est-à-dire une société qui reconnaisse à chaque personne des droits humains inaliénables et universels- civils, politiques, économiques, sociaux, culturels

qui s'opposent à toute logique d'exclusion et d'injustice sociale, qui garantissent et défendent la participation sociale de chacune et chacun, quelles que soient ses capacités. Il s'agit d'affirmer que chaque personne a sa place doit respecter celle des autres. En matière de droit à l'éducation, les enfants et les jeunes en situation de handicap sont particulièrement concernés par cette école qui ne s'adapte pas. Il est temps de prendre les mesures nécessaires pour aller vers une éducation véritablement inclusive et émancipatrice, respectueuse des droits humains. Les enfants et jeunes en situation de handicap connaissent de nombreux décrochages et ruptures de parcours, dus à l'inadaptation de la pédagogie. Des moyens financiers et du personnel d'encadrement formé pour garantir la scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire. Il faut rendre accessibles tous les lieux d'accueil, d'activités et d'enseignement, mais également former et soutenir les professionnels de l'éducation et de l'enseignement. Il faut enfin soutenir des structures adaptées, car tous les enfants en situation de handicap ne peuvent intégrer une école dite « ordinaire ». matière de droit au travail et à la formation, notre pays connaît un terrible retard. Est-il concevable que, en Île-de-France, Pôle emploi ne dispose que d'une seule personne référente sur ces questions ? Pour favoriser l'accompagnement en milieu ordinaire,

En conclusion, la personne en situation de handicap est aujourd'hui considérée non pas comme un sujet de droit, mais comme une personne ayant des incapacités. C'est ce paradigme qu'il convient de changer en adaptant notre législation. Je terminerai en citant cette phrase de Gabriel Garcia Marquez : « J'ai appris qu'un homme n'a le droit d'en regarder un autre de haut que pour l'aider à se lever. Je souhaite, madame la secrétaire d'État, que vous entendiez, dans mon propos et lors du débat qui va suivre, les exigences des personnes en situation de handicap et que vous puissiez faire mieux dans les six mois à venir. Je souhaite enfin que ce débat permette de faire avancer les droits de ces millions de femmes et d'hommes qui n'aspirent qu'à une seule chose : le respect. La parole

Cet échange offre l'occasion d'examiner les recommandations du Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU (CDPH), qui a auditionné la France sur l'application de la convention relative aux droits des personnes handicapées ratifiée en 2010. Si nous ne partageons pas la vision caricaturale présentée par le CDPH sur les établissements français accompagnant des personnes en situation de handicap, certaines recommandations vont dans le bon sens renforcer l'accessibilité des maisons pour femmes handicapées victimes de violences, prévenir le risque de suicide des personnes autistes ou en situation de handicap psychique, limiter les disparités territoriales dans l'accès aux droits, notamment en matière d'accessibilité numérique. Plus largement, nous devons renforcer les dispositifs de protection des adultes vulnérables contre toute forme de maltraitance, allant de la négligence aux violences actives. D'après les estimations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), une personne âgée sur six a été victime de maltraitance dans son environnement, qu'il soit familial ou institutionnel.

verbales ou sexuelles. Les femmes en situation de handicap sont deux fois plus souvent agressées à domicile ou près de chez elles, souvent par une personne de leur entourage. Le rapport sénatorial de la délégation aux droits des femmes publié en octobre 2019 décrit une situation alarmante pour les femmes autistes, dont 90 % seraient victimes de violences sexuelles. L'accès aux soins des personnes autistes se révèle parfois difficile. D'après les experts, de nombreuses personnes autistes ou Asperger, en particulier des femmes, mettent en place un mécanisme de camouflage social pour des raisons d'acceptation sociale et professionnelle. Si cette stratégie de dissimulation leur permet de ne pas être identifiées comme des personnes autistes et ainsi d'éviter une forme de stigmatisation, cela se fait bien souvent au détriment de l'accompagnement et du soutien dont elles auraient besoin. Ce mécanisme d'adaptation, qui concerne davantage les femmes, expliquerait pourquoi les hommes sont trois à quatre fois plus nombreux à être diagnostiqués autistes. Il faudrait, pour renforcer l'accès aux soins de ces personnes, adapter les outils diagnostiques à l'existence d'une spécificité féminine de l'autisme et du syndrome d'Asperger, moins visible et moins détectée. Nous savons que les personnes autistes sont particulièrement vulnérables au harcèlement, à la dépression et au suicide. Selon une étude publiée en 2014, deux personnes autistes sur trois déclarent avoir envisagé de se suicider. Ces chiffres sont extrêmement préoccupants. C'est pourquoi l'accompagnement de ces personnes trop souvent isolées est indispensable. généralisation, annoncée par le Gouvernement, à la suite des Assises de la santé mentale et de la psychiatrie, du remboursement des consultations de psychologue ou de psychothérapeute. Il s'agit d'une avancée importante pour améliorer l'accès à la santé de nombreuses personnes vulnérables, dont celles qui sont atteintes d'un handicap.

d'État, que cela soit réellement le cas en 2021 ? Les droits des personnes handicapées sont-ils pleinement effectifs aujourd'hui ? Pour le Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU, qui a publié ses conclusions portant sur l'application par la France de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, il semblerait que non. ce rapport sévère et inquiétant, « le modèle du handicap basé sur les droits de l'homme n'a pas été intégré dans la législation ni la réglementation nationales », pas plus qu'il n'est « devenu partie intégrante de la conscience politique et professionnelle » en France. Malgré la devise « Liberté, Égalité, Fraternité » du pays dit des droits de l'homme, les personnes en situation de handicap sont laissées de côté, a affirmé Jonas Ruskus, De toute évidence, il y a eu des avancées ces dernières années, notamment pour inscrire la question du handicap à l'agenda politique et bâtir une société plus inclusive. Des progrès sont à noter. Depuis la grande loi sur le handicap de 2005, de nombreuses mesures ont été annoncées par les différents gouvernements. Je pense par exemple à la modification du code du travail obligeant les employeurs à prendre des mesures d'aménagement raisonnables et assimilant le refus d'obtempérer en la matière à une discrimination fondée sur le handicap. Je pense aussi à la loi d'orientation destinée à favoriser l'autonomie des personnes handicapées et à la stratégie pour l'emploi des personnes en situation de handicap. En mars dernier, contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a voté en faveur de la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés

Il y a aussi la cinquième branche de la sécurité sociale dédiée à la perte d'autonomie : confirmée dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, sa mise en place est toutefois inaboutie. Ces mesures vont dans le bon sens, mais ne constituent pas toujours des engagements forts ... Dans les faits, qu'en est-il réellement des droits des handicapés en matière d'éducation, de cadre de vie, d'accessibilité, de droit à la vie, d'égalité, de non-discrimination ou encore de participation à la vie politique et publique ? Le Comité onusien retient trois points de vigilance sur lesquels la France doit évoluer : le placement systématique en institution des personnes handicapées ; les traitements médicaux sous contrainte, notamment chez les personnes ayant un handicap psychosocial ; le dépistage génétique prénatal des déficiences foetales, des déficiences foetales, notamment de la trisomie 21, basé sur des stéréotypes négatifs à l'encontre des personnes handicapées et entraînant leur dévalorisation. Le rejet prénatal des personnes porteuses de trisomie 21 se poursuit tout au long de leur vie. C'est ainsi que le Comité onusien reproche à la France le départ de personnes handicapées vers la Belgique- elles sont contraintes de s'exiler, faute de solutions dans notre pays. Si nous n'accueillons pas pleinement la différence et la fragilité, alors les personnes handicapées n'auront jamais les mêmes droits que les autres. Elles ont besoin d'aide afin de prendre toute leur place dans la société. C'est une révolution culturelle qu'il faut mener pour faire émerger cette société plus inclusive et faire changer le regard sur le handicap. L'accueil de la fragilité est le premier critère de notre humanisation. Prenons l'exemple de l'école. Le droit à l'éducation est garanti par l'article 24 de la convention relative aux droits des personnes handicapées. L'école est essentielle pour les enfants : ils y sont instruits et y apprennent les règles de la vie en collectivité. Pourtant, de trop nombreux élèves ne sont plus accompagnés, faute de moyens financiers et d'une pénurie d'accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH)- je le constate dans mon département. L'ONU dénonce ainsi le manque d'aménagements raisonnables pour répondre aux exigences éducatives, particulièrement pour les enfants autistes. Le sujet de l'éducation est primordial, il faut agir en est de même concernant l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Aujourd'hui, le taux de chômage des actifs handicapés atteint 19 %. Les entreprises préfèrent payer une contribution plutôt que de respecter le quota ce n'est pas acceptable ! Nous devons favoriser la rencontre entre l'entreprise et la personne handicapée. Cela constitue bien souvent un choc positif pour l'entreprise, fabrique de la solidarité et accompagne les personnes handicapées vers l'indépendance.

Les démarches auprès des administrations sont parfois complexes et des difficultés existent pour certains dossiers. La non-fourniture d'un document ou l'incompréhension sur une demande peut entraîner des suspensions de droits pour les personnes handicapées.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, 12 millions de personnes sont touchées par un handicap en France. La loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a permis de réelles avancées,

De même, l'ensemble des collectivités locales devraient être accompagnées et bénéficier d'un vaste plan leur permettant de concrétiser plus rapidement la mise en accessibilité de leurs structures, transports ou services.

Plutôt que de garantir un nombre de places suffisant, vous développez des services annexes comme la RAPT, le PAG et maintenant le PCPE, autant d'acronymes qui sont incompréhensibles pour les familles, mais qui ne masquent pas l'absence criante de structures adaptées

», renforcer la formation des enseignants et élaborer un véritable partenariat entre l'école et le médico-social. Pour conclure, permettez-moi de revenir sur un sujet d'actualité

nous sommes nombreux ici à le dire, comme les personnes concernées et les acteurs de l'accompagnement du handicap. Cette légitime revendication doit être entendue. Soyez sûre, madame la secrétaire d'État, que la mobilisation ne faiblira pas sur ce sujet

emploi, culture, sport. Je n'ai pu esquisser ici que quelques-unes des pistes de travail sur lesquelles nous souhaitons que tout le monde se penche. La

le débat qui nous est proposé aujourd'hui sur l'initiative de nos collègues du groupe CRCE, que je remercie, porte non seulement le droit des personnes en situation de handicap, et donc l'accès à leurs droits, mais également le soutien que nous devons à ceux qui, proches aidants, apportent une assistance essentielle aux personnes malades, âgées ou handicapées. En 2020, la Conférence nationale du handicap a permis la signature d'un accord de méthode sur le pilotage et le fonctionnement des MDPH. Il engage l'État et les départements vers une simplification de l'accès aux droits de façon équitable sur l'ensemble du territoire. Plus récemment, la feuille de route MDPH 2022 a énoncé des objectifs similaires, à savoir un accès aux droits plus simple, plus efficace et plus équitable sur l'ensemble du territoire.

Madame la secrétaire d'État, pouvez-vous nous dire si la moyenne de ces délais s'améliore ? Si oui, de combien ? Surtout, pouvez-vous, dans votre réponse, distinguer le délai moyen de traitement des premières demandes et des demandes de renouvellement ? Dans un souci d'amélioration du service rendu, tant en termes d'efficacité que d'égalité des territoires, quels leviers pourrait-on actionner afin que les départements puissent améliorer ces délais ? Hier se déroulait la journée nationale des aidants.

si le besoin de répit a été identifié lors de l'examen ou du réexamen de la prestation. Si le besoin apparaît en dehors de ces périodes et que le besoin est soudain, la prise en charge devient plus difficile. En 2015, soit dix ans plus tard, la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement réformait l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et consacrait, à la différence de la PCH, un module en faveur du répit d'environ 500 euros par an, permettant le financement d'une solution de répit. Cette enveloppe sanctuarisée montre l'évolution de la place de l'aidance dans nos politiques publiques. J'ajoute toutefois que, juridiquement, rien ne s'oppose au financement du répit sur le volet relatif à l'aide humaine du plan APA, lorsque ce volet n'est pas saturé et que le département y consent. Si je fais ce parallèle, madame la secrétaire d'État, c'est que le champ des personnes handicapées et des personnes âgées relève d'une approche similaire, celle de l'autonomie.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a permis de réaffirmer le droit à l'éducation des personnes en situation de handicap. Le Le texte pose les principes de l'école inclusive et prévoit que tout enfant ou adolescent en situation de handicap est de droit inscrit dans l'établissement d'enseignement le plus proche de son domicile. En 2010, la France ratifiait la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et réaffirmait ainsi sur la scène internationale son engagement à protéger les personnes en situation de handicap et à leur garantir

notamment la présence de structures qui, selon lui, perpétuent la stigmatisation et l'exclusion des enfants en situation de handicap, désignant les IME et les ULIS. Cette préoccupation, qui ne doit pas remettre en cause les bénéfices de ces structures, doit en revanche nous inviter à faire preuve de vigilance et à privilégier le milieu scolaire ouvert chaque fois que cela est possible. est insuffisant, alors qu'il est pourtant nécessaire pour permettre, en particulier aux enfants atteints d'autisme et de trisomie, de satisfaire les exigences académiques requises. Le Comité déplore aussi la faiblesse de la part des personnes en situation de handicap qui accèdent à l'enseignement supérieur. Au cours de l'année universitaire 2020-2021, 40 000 personnes en situation de handicap suivaient une formation d'enseignement supérieur c'est certes 14 000 personnes de plus que l'année précédente, mais cela ne représente qu'un étudiant sur cinquante, alors que plus d'un Français sur six est en situation de handicap. Le Comité constate également une insuffisance de données statistiques sur la scolarisation des enfants en situation de handicap résidant dans les territoires ultramarins. insuffisantes pour certaines populations malheureusement marginalisées : les Roms, les demandeurs d'asile ou encore les réfugiés. Autre point : le Comité reproche à la France de n'avoir pas pu fournir des équipements satisfaisants aux enfants en situation de handicap lors de la crise sanitaire, en particulier aux enfants malentendants. La pandémie a, on le sait, contribué à aggraver les disparités dans l'éducation et l'absence d'équipements adaptés a constitué un obstacle de plus à l'inclusion. Enfin, le Comité a jugé insuffisant l'enseignement dispensé en langue des signes, ainsi que celui de la langue des signes elle-même. Il déplore encore l'absence d'usage et d'enseignement du braille.

sont pourtant un maillon essentiel de la scolarisation de ces élèves grâce à leur travail d'accompagnement et de socialisation. Les accompagnants décrivent des conditions de travail difficiles, accentuées par la mise en place des pôles inclusifs d'accompagnement localisés. Ce nouveau dispositif d'organisation du travail des AESH a pu avoir pour effet de confier à l'accompagnant un groupe d'élèves trop nombreux, ne lui permettant plus d'assurer son travail dans les meilleures Hier encore, à Lyon, dans mon département, 2 000 professionnels du secteur médico-social manifestaient devant la préfecture pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail et le manque de personnel qualifié et pour demander l'extension du Ségur de la santé aux établissements médico-sociaux. Le bilan n'est cependant pas entièrement négatif : des progrès ont été réalisés, notamment, comme je l'ai évoqué, en termes d'accès à l'enseignement supérieur, mais la situation demeure perfectible. La semaine prochaine, le Sénat examinera en deuxième lecture la question de la prise en compte des revenus du conjoint dans le calcul de l'allocation aux adultes handicapés. Je forme le voeu que le Sénat fasse, de nouveau, le choix de l'extension des droits des personnes en situation de handicap.

Le respect des droits passe inévitablement par une bonne prise en charge des personnes et donc par la garantie d'un accompagnement adapté et qualifié. Les professionnels qui ont pour mission de « prendre soin » doivent eux-mêmes se sentir bien dans leur métier. Or l'actualité et les sollicitations dont nous faisons l'objet dans nos départements nous interpellent. Ce mardi 5 octobre, à l'appel d'organisations syndicales et de jeunesse s'est tenue une journée de manifestation interprofessionnelle. Les professionnels du secteur médico-social étaient en première ligne. Hier, 6 octobre, à l'occasion de la journée nationale des aidants, des mobilisations ont eu lieu dans toute la France autour des métiers du soin et de l'accompagnement des personnes dépendantes. Les professionnels du secteur du handicap, les personnes en situation de handicap et leurs familles étaient nombreux pour dire leur impatience face aux tensions majeures et au risque que la pénurie de main-d'oeuvre fait courir aux personnes accompagnées. Tous tirent la sonnette d'alarme sur le manque de moyens, qui met en péril les métiers du « prendre soin » et en danger le respect des droits des personnes en situation de handicap. Problèmes de recrutement, manque de reconnaissance, épuisement des personnels dans le secteur médico-social, notamment celui du handicap, les démissions et l'absentéisme sont en augmentation. Le Ségur a créé une concurrence entre les structures selon leur statut et nous constatons un mouvement de fuite des agents vers celles où ils sont désormais mieux rémunérés. Le Gouvernement a proposé une hausse de salaire de 183 euros net par mois aux personnels des Ehpad et des hôpitaux publics, mais il a écarté ceux du secteur privé non lucratif du handicap. L'accord résultant de la mission Laforcade, censé corriger les inégalités, a provoqué de nouvelles désillusions au sein des associations gestionnaires d'établissements médico-sociaux pour personnes handicapées, en créant de nouvelles incohérences, cette fois-ci entre professionnels d'un même établissement. La question de la juste valorisation salariale pour l'ensemble des professionnels n'est pas le seul point de tension du secteur. Promotion des métiers, politique de formation, évolution de carrière, qualité de vie au travail : la question de l'attractivité du secteur doit être retravaillée dans son ensemble pour une prise en charge de qualité des personnes en situation de handicap. Cette pénurie a des effets délétères sur le bien-être des usagers, principalement dans les établissements médicalisés, qui ont dû mettre en place des fonctionnements dégradés. Les professionnels du secteur, les associations et les familles des personnes en situation de handicap nous alertent sur le nombre croissant de défauts de soins observés ces derniers mois.

C'est là une atteinte à leur dignité. Ces personnes deviennent alors des objets de soins. Le recours à des intérimaires, à des bénévoles ou à des retraités manquant souvent de formation ne constitue pas une solution. Certaines structures se voient aujourd'hui contraintes de fermer des services et de limiter les accueils de jour. Nous sommes surpris de constater que l'avant-projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 ne prévoie pas les compensations financières liées aux revalorisations salariales des professionnels de l'accompagnement. Le projet de loi relatif à l'autonomie aurait pu être l'occasion de répondre à ces inquiétudes et de remettre à plat la prise en charge du handicap dans notre pays, mais nous savons désormais qu'il ne verra pas le jour durant ce quinquennat

le groupe CRCE a souhaité inscrire à l'ordre du jour de nos travaux un débat sur les droits des personnes en situation de handicap. Je tiens à saluer cette initiative et à rappeler la nécessité pour notre assemblée de s'exprimer régulièrement sur cette question. Nous le devons bien sûr aux 12 millions de Français touchés par un handicap, particulièrement aux 9 millions d'entre eux dont le handicap est invisible. nécessaire aussi afin de mesurer le chemin parcouru depuis l'adoption en 2005 de la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et depuis l'entrée en vigueur en 2008 de la convention relative aux droits des personnes handicapées. Ce débat est également l'occasion d'évaluer la politique du Gouvernement en la matière et les efforts consentis pour assurer l'effectivité et le respect des droits des personnes en situation de handicap. Ces droits, quels sont-ils ? C'est le droit de vivre, de se former, de travailler, d'avoir une vie intime et personnelle, de se déplacer en sécurité, de s'épanouir. Cela semble une évidence, et pourtant C'est aussi le droit de bénéficier d'une compensation financière pour faire face à des situations de vie souvent difficiles. Je pense à la prestation de compensation du handicap et à l'allocation aux adultes handicapés- cette dernière a d'ailleurs été revalorisée à deux reprises depuis le début du quinquennat. Avec un budget annuel de 51 milliards d'euros, soit 2,2 % du PIB, la France figure à la troisième place des pays européens en termes de financement des politiques consacrées au handicap. Cependant, beaucoup reste à faire. La Défenseure des droits en a fait le constat il y a quelques mois dans un rapport sur la mise en oeuvre par la France de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Le Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies s'en est d'ailleurs ému. S'il a salué l'ambition de la stratégie nationale pour l'autisme ou la feuille de route pour la santé sexuelle des personnes handicapées, il a critiqué une approche jugée trop médicale et souligné l'urgence d'accroître nos efforts pour lutter contre la stigmatisation. Si beaucoup reste à faire, il est utile, je pense, de rappeler l'ampleur du travail accompli depuis le début du quinquennat : 400 000 élèves en situation de handicap étaient scolarisés à la rentrée 2021, soit près de 20 % de plus qu'en 2017. Nous agissons en faveur de leur droit à l'éducation. Nous agissons aussi en faveur de leur droit à une inclusion totale dans leur lieu de vie, grâce à la création des communautés 360, ou dans leur vie professionnelle. Le nombre d'apprentis en situation de handicap a ainsi bondi de 3 500 en 2019 à près de 6 000 en 2020. Depuis janvier 2021, 15 000 recrutements, dont les deux tiers en ont été réalisés dans le cadre du plan de relance, au titre de l'aide à la mobilisation des employeurs pour l'embauche des travailleurs handicapés. Nous agissons enfin pour leur droit à la protection. Je pense notamment aux projets pilotes en Gironde et en Loire-Atlantique lancés en octobre 2020 pour le soutien et l'accompagnement des femmes en situation de handicap victimes de violences conjugales. J'évoquerai ici la situation particulière des outre-mer, où les besoins sont plus nombreux qu'ailleurs et où les retards en matière de politique du handicap sont réels. Une enquête menée par la Drees et l'Insee en 2019

L'écart est encore plus frappant si l'on compare les chiffres de la population âgée. Ainsi, 21 % des personnes âgées de 55 ans ou plus sont handicapées en Guadeloupe, en Guyane et à La Réunion ; ils sont 24 % en Martinique et à Mayotte, contre 16 % dans l'Hexagone. À cet écart, qui exige des moyens adaptés, s'ajoute le retard de prise en charge des personnes handicapées. Dans un rapport de septembre 2019 consacré à l'accès aux droits dans les outre-mer, la Défenseure des droits notait ainsi que « les insuffisances des dispositifs sanitaires et les inégalités d'accès à la santé y favorisent le renoncement aux soins, ainsi que les discriminations envers les personnes en mauvaise santé, âgées ou en situation de handicap Ce constat est particulièrement vrai en ce qui concerne la scolarisation et l'accompagnement des plus jeunes. La détection des situations de handicap, faute de moyens suffisants, y est ainsi plus difficile qu'ailleurs.

à être temporaires, s'inscrivent parfois dans la durée. La consultation sur les discriminations, lancée en avril dernier pour recueillir les propositions des citoyens, et la plateforme de signalement et d'accompagnement des victimes ou témoins de discriminations

avec le débat sur le thème : « Les droits des personnes en situation de handicap sont-ils effectifs et respectés ? »

le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, garantir l'accès à l'éducation et à une formation qualifiante, c'est préparer l'avenir de nos enfants, tant socialement que professionnellement. Le 4 septembre dernier, des milliers d'enfants ont rejoint le chemin de l'école pour la rentrée scolaire. Malheureusement, certains d'entre eux, en situation de handicap, n'ont pas eu cette chance. Aujourd'hui, entre 8 000 et 11 000 enfants en situation de handicap- la majorité présente un handicap cognitif ou intellectuel -restent sans solution. De fait, certains enfants sont exclus de l'école de la République. Cette absence de solution hypothèque leur avenir et met les familles en difficulté. Le nombre limité d'auxiliaires de vie scolaire, d'assistants d'élèves en situation de handicap et d'unités localisées pour l'inclusion scolaire complique la scolarisation. Les enfants présentant un handicap mental sont particulièrement touchés. Or les conséquences du déficit de scolarisation sont lourdes : retards d'apprentissage, manque de socialisation, difficultés d'intégration et autant de potentiels ignorés. Cette inégalité des interrogations. Stephen Hawking aurait-il été le physicien et le théoricien que nous connaissons s'il avait été français et atteint d'un handicap dès la naissance ? Quelles auraient été ses chances de devenir le chercheur et l'intellectuel qu'il a été ?

Les données dont nous disposons confirment ce diagnostic : l'insuffisante scolarisation des personnes handicapées induit un faible niveau de formation, qui nuit à leur intégration sociale. On constate que le niveau de handicap décroît tendanciellement avec le niveau de diplôme. En d'autres termes, plus le handicap d'un individu est important, plus son niveau de diplôme est bas.

dont nous savons, madame la secrétaire d'État, que vous mesurez pleinement l'ampleur. La France compte aujourd'hui 3,5 millions de personnes en situation de handicap, dont 700 000 en situation de handicap mental. Quelles solutions comptez-vous apporter

le sexe », conformément à l'article 16 de la convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée par les Nations unies en 2006 et signée par la France. pourtant que ce droit à la protection contre les violences sexuelles n'est pas correctement assuré, en particulier dans les institutions accueillant des mineurs en situation de handicap.

presque systématique, pour les jeunes filles atteintes de troubles autistiques : 90 % d'entre elles subissent des violences sexuelles et 31 % subissent un viol avant l'âge de 9 ans, en raison de leur immense vulnérabilité. Face à ces fléaux, nous proposions quelques pistes pour améliorer la protection des enfants handicapés : renforcer les contrôles des nombreux intervenants, d'une part, développer les mesures de prévention, d'autre part. Le premier moyen de protéger les enfants est de contrôler qu'ils ne sont pas exposés à des adultes auteurs d'infractions sexuelles. C'est le but du Nous notions, en 2019, que ce fichier était méconnu des directions d'établissements accueillant des enfants handicapés et que sa consultation n'était pas systématique, faute d'habilitation des services recruteurs. En février 2020, le Gouvernement a mesuré la marge de progrès pour faire du Fijais le point nodal de la lutte contre le renouvellement des infractions. secrétaire d'État, sur les résultats de l'audit effectué par le ministère de la justice : des procédures de téléconsultation du Fijais et du bulletin n° 2 du casier judiciaire sont-elles mises en place pour les établissements médico-sociaux, à l'instar de ce qui se pratique dans les centres de loisirs ?

les mesures de prévention mises en oeuvre, par l'absence totale de procédure et même de réflexion sur les pratiques professionnelles des deux grands réseaux associatifs gestionnaires d'établissements auditionnés. Ces préoccupations semblaient totalement hors de leurs radars. Là encore, le plan du Gouvernement prévoyait « dès 2020 des formations communes pour renforcer la coopération entre professionnels sur les violences intrafamiliales ». En revanche, aucune stratégie n'a été définie pour accroître le repérage et le signalement des violences commises dans les établissements. Il nous semble primordial que ces enjeux soient inclus dans les modules de formation initiale et continue des professionnels. C'est ainsi que nous avancerons vers un meilleur droit à

madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, en 2021, la place des Français en situation de handicap demeure un enjeu majeur. Près de 12 millions de Français sont actuellement touchés par un handicap et souffrent d'une incapacité ou d'une limitation d'activité. Certes, les politiques publiques en faveur de l'intégration des personnes en situation de handicap ont été renforcées ces dernières années. Je pense bien sûr à la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, L'objectif de favoriser l'intégration des personnes handicapées et leur participation à la vie sociale demeure tout aussi important. Pour atteindre cet objectif, la loi privilégiait les éléments essentiels d'une vie normale à laquelle chacun aspire l'accès aux lieux publics, aux transports en commun, à un logement, ainsi que l'obtention d'un travail adapté. Pourtant, quinze ans après son entrée en vigueur, l'effectivité de cette loi reste incertaine. ans après la loi pour l'égalité des droits et des chances, 18 % des personnes souffrant de handicap sont au chômage, soit près du double de la moyenne nationale. 67 % des personnes souffrant de handicap font face à un manque d'accessibilité des lieux publics et déclarent rencontrer des difficultés pour se déplacer. Dans cette optique, le 14 septembre dernier, le Comité des Nations unies pour les droits des personnes handicapées relevait les limites de la loi pour l'égalité des droits et des chances Le Comité regrette par ailleurs que la loi de 2005 définisse un « modèle de prise en charge médico-sociale » favorisant l'institutionnalisation systématique sur la base du handicap. Les Nations unies ont, par conséquent, recommandé à la France de mettre en oeuvre des stratégies afin d'éliminer les représentations négatives ou dévalorisantes des personnes handicapées. L'ONU a par ailleurs encouragé la France à renforcer les mécanismes tels que la surveillance indépendante et le contrôle judiciaire afin de prévenir toutes les formes de mauvais traitements et de protéger de la surmédication les enfants handicapés placés en institution. Nos concitoyens en situation de handicap ont en principe les mêmes droits que le reste de la société. En pratique, l'application de ces droits reste souvent parcellaire. L'exemple de aux adultes handicapés illustre cette inégalité des droits. De nombreuses propositions de loi ont été déposées afin de désindexer l'AAH des revenus du conjoint et du foyer, mais le Gouvernement s'y est malheureusement encore opposé. Difficultés de niveau de vie, impossibilité d'obtenir l'AAH en deçà d'un certain degré de handicap, baisse de l'AAH de la personne en situation de handicap au fur et à mesure qu'augmentent les revenus du conjoint valide, impossibilité d'acquisitions immobilières : les problématiques posées par l'AAH sont multiples et reflètent la situation à laquelle se heurtent encore nombre de nos compatriotes en situation de handicap. L'ONU invite d'ailleurs le Gouvernement à réformer le règlement de l'AAH en ce sens. Nous le constatons encore et encore, la personne handicapée est considérée comme une personne souffrant d'incapacités avant d'être considérée comme un sujet de droit. Il nous revient dorénavant de changer ce paradigme, pour peu que nous voulions réellement que notre pays franchisse une étape importante pour l'inclusion des personnes handicapées. La parole est

En quatre ans, beaucoup a déjà été accompli pour rendre notre société toujours plus inclusive et pour faire toute leur place aux 12 millions de personnes en situation de handicap et à leurs 8 millions d'aidants.

indemnisé depuis octobre 2020, et nous investissons dans le développement de solutions de répit. Nous disposons ainsi d'une feuille de route ambitieuse pour la dernière dernière partie du mandat, établie en concertation avec les personnes en situation de handicap, les associations, les collectivités locales et, bien sûr, la société civile et dont les objectifs ont été renforcés par le contexte de la crise sanitaire, économique et sociale. Dans le champ du handicap, quatre réformes prioritaires ont été intégrées au dispositif gouvernemental : elles visent à simplifier l'accès aux droits pour les personnes handicapées, permettre une intervention précoce auprès des enfants souffrant de troubles du neuro-développement, à offrir une scolarité inclusive et adaptée à tous les enfants handicapés et, enfin, à mieux accompagner les aidants. Je vais à présent vous présenter les deux réformes dont le secrétariat d'État assure le pilotage en vous faisant part à chaque fois de leur état d'avancement et de l'ambition que nous portons d'ici la fin du mandat, chère Sophie Cluzel. première réforme prioritaire porte sur la simplification de l'accès aux droits des personnes handicapées. Depuis le début du quinquennat, le Gouvernement conduit une politique volontariste pour simplifier durablement l'accès aux droits des personnes en situation de handicap et assurer une équité territoriale, quel que soit le lieu de résidence des personnes concernées. Nous avons fait le choix de mobiliser tous les leviers réglementaires et budgétaires pour permettre aux MDPH d'accélérer le traitement des dossiers afin que nos concitoyens bénéficient de leurs droits sans avoir à multiplier les démarches. C'est la logique qui a sous-tendu la création, au début de l'année 2019, de droits sans limitation de durée pour les personnes dont le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement, le passage de six à douze mois de la validité des certificats médicaux, la simplification des formulaires de demande ou le déploiement d'un système d'information harmonisé pour près de 99 MDPH. Nous menons cette action en lien étroit avec les conseils départementaux dans le cadre de la Conférence nationale du handicap. Le 11 février 2020, un accord de méthode inédit a été signé entre l'État et l'Assemblée des départements de France pour optimiser de façon significative, en deux ans, le pilotage et le fonctionnement des MDPH. Après des années de stagnation, l'État mobilise désormais d'importants moyens financiers

et de l'activité des MDPH afin de soutenir l'équité de la réponse. Par ailleurs, pour soutenir les départements, la CNSA a mis en place une équipe de sept personnes afin d'épauler les MDPH sur le terrain et améliorer leur processus de traitement et leur pilotage. Il s'agit de réduire le stock des dossiers. Enfin, pour permettre en toute transparence à chaque citoyen de suivre les avancées et de s'assurer de l'équité territoriale de notre action, nous avons créé, avec Dominique Bussereau, le baromètre des MDPH. Il s'agit d'un tableau de bord de l'activité des 104 MDPH, qui permet chaque trimestre la progression des différents chantiers et de favoriser une dynamique positive entre les territoires. L'ensemble de nos actions permet aujourd'hui de disposer d'indicateurs très

seconde réforme prioritaire vise à permettre une intervention précoce auprès des enfants atteints de troubles du neuro-développement. Chaque année, 35 000 enfants en moyenne naissent en France avec un trouble du neuro-développement. Ils sont diagnostiqués en moyenne vers l'âge de 6 ou 7 ans, alors même qu'il est possible de repérer ces troubles plus précocement. L'enjeu est ainsi d'agir tôt, alors que l'enfant bénéficie encore d'une grande plasticité cérébrale permettant d'améliorer son développement. Le forfait « intervention précoce » est l'une des mesures phares de la Stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neuro-développement pour la période 2018-2022. L'objectif de ce nouveau dispositif est d'identifier le plus tôt possible ces troubles afin de mettre en place pour les enfants de 0 à 7 ans une intervention adaptée afin de favoriser leur développement et de

capables de proposer aux familles, dès les premiers signes d'alerte, des interventions adaptées ou bien de les orienter vers les professionnels libéraux respectant les recommandations de bonnes pratiques, avec lesquels elles auront passé un contrat. L'intégralité du parcours est évidemment pris en charge par l'assurance maladie. Un forfait pendant 24 mois afin de rémunérer les interventions de psychologues, ergothérapeutes, psychomotriciens exerçant en libéral, dont les bilans n'étaient jusqu'alors pas remboursés. Cela représente pour les familles une dépense évitée de 1 500 euros en moyenne. À ce jour, 63 plateformes sont d'ores et déjà en place et 15 plateformes supplémentaires seront ouvertes avant l'été. Elles auront permis de repérer plus précocement 6 800 enfants et de déclencher 3 807 forfaits de bilan et d'intervention précoce. D'ici 2022,

les premières plateformes dédiées aux enfants de 7 ans à 12 ans présentant des troubles du neurodéveloppement seront également mises en place dès 2021. Vous pouvez constater que cette réforme change profondément la vie des enfants diagnostiqués et de leurs familles. Il nous faut continuer dans cette voie en mobilisant encore davantage les professionnels de la petite enfance, les médecins généraux et les pédiatres, en lien avec la Caisse nationale

des droits et le meilleur accompagnement possible dans un projet de société toujours plus inclusive. Madame

l'initiative de mon groupe, Les Indépendants - République et Territoires, le Sénat a créé en mai dernier une mission d'information sur le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. Présidée par notre collègue Sabine Van Heghe, que je tiens ici à saluer et à remercier pour sa présidence efficace et attentive, notre mission a travaillé dans une ambiance studieuse et confiante, qui est la marque de fabrique du Sénat. du Sénat. Le harcèlement scolaire et son développement dans le cyberespace constituent une préoccupation très largement partagée, qui nous concerne tous. En effet, il s'agit d'un fléau qui, surtout dans sa dimension « cyber sape insidieusement les fondements du vivre ensemble. Nous devons donc décréter la mobilisation générale pour mieux prévenir, détecter et traiter, afin de suivre efficacement les victimes et de disposer d'un réel suivi des harceleurs.

Mais, et ce sera mon second point, nous avons une ardente obligation de tout faire pour endiguer et éradiquer ces ferments de haine. La mobilisation générale que nous préconisons doit devenir sans tarder une grande cause nationale, et nous comptons sur votre implication, madame la secrétaire d'État, pour faire aboutir cette recommandation. Je commencerai mon propos en revenant sur le constat actuel, très largement partagé, concernant l'acuité de ce fléau du harcèlement. Le harcèlement scolaire- chacun le voit dans son environnement personnel ou familial -est un drame individuel, mais aussi collectif. Il n'épargne personne, aucun milieu, aucun établissement, d'autant plus que les réseaux sociaux, par leur puissance, leur anonymat, leur viralité et leur évolution permanente en démultiplient les effets dramatiques. Se crée ainsi, pour reprendre une expression largement répandue parmi les acteurs du monde de l'éducation, un « continuum de violence » entre l'école et la sphère privée. Les chiffres qui figurent dans notre rapport le montrent en détail : près d'un élève sur dix en est victime ; dans sa version « cyber », il se concentre surtout sur les jeunes filles et stigmatise toutes les différences.

Il faut ainsi saluer et reconnaître à sa juste mesure tout ce travail. C'est en réalité la prise en charge du « dernier kilomètre » qui fait souvent défaut. Elle suppose une capacité d'écoute qui est propre à des adultes formés pour cela, une stabilité des équipes, une libération de la parole des enfants, un suivi de la victime et l'adoption de sanctions éducatives contre les harceleurs. Nous devons également relever un double défi. D'une part, la panoplie actuelle des instruments de lutte contre le harcèlement est assez, voire paradoxalement trop étendue. Des numéros d'appel, ainsi qu'un site public dédié existent, sans oublier un concours national et une journée annuelle de sensibilisation, le dispositif des « élèves ambassadeurs » ou les opérations locales de sensibilisation. Mais, en réalité, nombre de ces outils sont mal connus ou insuffisamment utilisés. D'autre part, il nous semble que l'arsenal juridique est, pour une large part, insuffisant face au cyberharcèlement. En droit français, le harcèlement est déjà pénalement réprimé, notamment lorsque les actes sont effectués en meute.

que des messageries privées protégées par le secret des correspondances, et le siège de ces réseaux n'est pas situé en France ni même en Europe. Madame la secrétaire d'État, nous comptons sur l'engagement déterminé du Gouvernement, car une action juridique solide et efficace ne peut se concevoir que dans un cadre européen, voire international. De ce fait, et c'est mon second point, notre mission d'information a pour objet très précis d'accélérer la prise de conscience et la mise en place de nouvelles réponses mieux adaptées à l'environnement « cyber

Quel effet a eu le confinement sur le harcèlement et le cyberharcèlement ? Les premières indications accréditent l'idée d'une stagnation du harcèlement classique et, à l'inverse, d'une augmentation du cyberharcèlement,

Les élèves harcelés ne doivent faire aucun effort de mémorisation au moment où ils estiment nécessaire de recourir à ces numéros. En outre, nous avons regardé les solutions mises en place dans d'autres pays comparables au nôtre, qui ont fait la preuve de leur efficacité. Comme dans les pays scandinaves, il faut promouvoir le maintien ou la construction d'un climat scolaire de qualité autour de la notion du vivre ensemble. Il y a matière à faire évoluer la formation initiale et continue, non seulement des enseignants, mais aussi, plus globalement, de toute la communauté éducative. Surtout, chaque enfant doit connaître précisément ses droits et ses devoirs. Un document d'information, dont le contenu sera annexé au projet d'établissement, doit être distribué chaque année au moment de la rentrée pour rappeler le droit existant, les numéros d'appel et les sanctions encourues. Une autre de nos priorités est de développer notre capacité à détecter rapidement une situation de harcèlement et, notamment, à repérer les signaux dits « faibles ». Il s'agit, par exemple, des élèves qui, sans raison apparente, durant plusieurs jours, ne terminent pas leur repas de midi à la cantine. L'enfant ne doit pas avoir peur d'aller en parler avec des adultes de confiance, que ce soit l'enseignant, le conseiller principal d'éducation (CPE), l'assistant d'éducation, l'infirmière scolaire ou le personnel de la cantine.

il faut évidemment traiter systématiquement, et sans délai, tous les cas de harcèlement. Les élèves et leurs parents doivent bien savoir qu'aucun fait ne restera sans sanction, car le harcèlement est illégal. Toutes les victimes doivent être aidées. Dans une visée éducative, il faut concilier justice « restaurative », en généralisant les stages et les travaux d'intérêt général, et sanction des harceleurs. Il faut aussi éviter que, comme trop souvent, ce soit l'élève harcelé qui doive quitter l'établissement et qui soit ainsi victime d'une double peine. Nous demandons aussi que les suites réservées à ces cas de harcèlement soient systématiquement examinées par le conseil d'administration de l'établissement, ce qui n'est que trop rarement le cas. Ce traitement systématique doit permettre à chaque élève, qu'il soit victime, harceleur ou même témoin, de comprendre que le harcèlement n'est pas toléré, et que telle ou telle moquerie, tel ou tel geste, même pour jouer ou plaisanter, constitue pour l'enfant qui le subit un fait de harcèlement. En effet, à de nombreuses reprises, il nous est apparu que le harceleur, le témoin et même la victime n'arrivaient pas à percevoir ce qui caractérise pourtant un harcèlement. Enfin, à l'heure des réseaux sociaux, il faut que vous nous aidiez à gagner la course contre la montre engagée en matière de lutte contre la propagation des actes de malveillance sur internet. Bref, il faut que les réseaux soient enfin proactifs. Nos auditions le prouvent bien, il leur reste encore beaucoup de chemin à parcourir.

d'une part, la mise en place de pour vérifier que les objectifs assignés aux réseaux sociaux en matière de suppression des contenus litigieux sont bien atteints ; d'autre part, le développement du pour favoriser la dissuasion par la publicité, en stigmatisant les mauvais élèves du cyberespace.

dès 2022 ou 2023 notre prochaine grande cause nationale. Dans cette attente, je vous remercie, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, de votre attention. La

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, l'enfance est de ces temps fragiles que le regret ignore et la souffrance effleure. Elle est l'aube des promesses, la démonstration, parfois trompeuse, mais toujours nécessaire, de l'innocence, de l'illusion. Cette enfance est bercée des devoirs bénéfiques de l'apprentissage du destin d'adulte et de la vie collective. L'école, quant à elle, est d'abord le balbutiement de la conscience d'autrui, le lieu de l'apprentissage, du savoir, le temple de l'instruction. Cette école permet à nos enfants de grandir et de s'épanouir, tant sur le plan personnel, en tant qu'individus, que collectif : ils deviennent ainsi des citoyens vertueux, ouverts aux autres et sur le monde. Pour tous nos jeunes compatriotes, voilà ce que devrait être l'enfance et ce que devrait être l'école. Je viens en vérité de vous décrire un idéal déchu, tant cette école est peu à peu devenue pour beaucoup de nos enfants, et par le seul fait du harcèlement, un lieu de souffrance, de mal-être et de violence. Le développement du cyberharcèlement a accentué ce phénomène, en instaurant un continuum pervers de violence invisible, qui va bien au-delà du portail des établissements. Le rapport de notre mission d'information a mis en exergue l'ampleur du phénomène. trente-cinq recommandations, ce rapport est déjà plus qu'un thermomètre et bien davantage qu'une boussole, mais c'est d'un électrochoc que nous avons besoin. C'est devant les réalités vertigineuses du mal-être des jeunes Français, encore illustrées par le suicide d'une élève de 12 ans dans le Pas-de-Calais, il y a tout juste une semaine, que nous prenons conscience du déni dans lequel nous étions plongés. Alors que 700 000 élèves, soit deux à trois enfants par classe en moyenne, sont concernés par le harcèlement, alors qu'une victime sur quatre a déjà songé au suicide, alors que la médecine scolaire ne met à la disposition des établissements qu'un professionnel pour 12 000 élèves,

Alors que faire ? Détecter ? Oui. Traiter ? Bien sûr. Sanctionner ? Si nécessaire. Le mot clé est réactivité, car notre ennemi est le temps le temps de la compréhension, de la réaction, du témoignage, ce temps qui écrase, dilue et parasite l'action. La réactivité passe d'abord par l'action du témoin. Le ou les témoins, ce sont d'abord les élèves eux-mêmes, ce public des harceleurs, ces camarades des harcelés, qui constatent la souffrance de leurs pairs, mais qui ne donnent pas l'alarme de peur d'être perçus comme des délateurs. Construire une culture de la vigilance, c'est d'abord briser l'omerta de ceux qui voient ; c'est inverser la charge de l'anonymat qui déresponsabilise aujourd'hui l'agresseur, alors qu'il devrait protéger et libérer le lanceur d'alerte. Nous devons offrir aux témoins la faculté de sonner l'alarme sans risquer de représailles. Appuyons-nous sur les solutions existantes. Je citerai à cet égard l'application The Sorority, qui permet le renseignement instantané des signaux faibles en matière de lutte contre les violences conjugales. Pourquoi ne pas envisager la territorialisation d'un outil numérique similaire dans chaque établissement ? Chaque école, collège ou lycée disposerait ainsi d'un signal d'alarme efficace. Pourquoi ne pas recourir aux applications existantes du type OSE ou Pronote, qui relient parents, professeurs et élèves, et y adjoindre un lanceur d'alerte anonyme ? Une fois l'alerte donnée, c'est au système éducatif, parents compris, d'intervenir pour couper net les racines du harcèlement. La clé, disais-je, c'est la réactivité, et cela vaut bien sûr pour le cyberharcèlement, tant l'internet constitue l'espace des flux où se répand l'information à une rapidité parfois mortelle. À la dictature de la vitesse et de la réputation, opposons un principe de précaution qui imposerait aux réseaux sociaux de bloquer un contenu, dès lors qu'il met en péril l'intégrité d'un élève.

Oui, mes chers collègues, il est impérieux de s'attaquer à la racine du mal, car le sacrifice de l'enfance est aussi celui du développement personnel et de la vie collective. C'est en pensant à Fénelon que j'ai été amenée à cette conclusion : « Les premières années de l'enfance sont les plus précieuses, elles décident du sort des autres. » La parole

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, à l'école, les vexations, les humiliations et, parfois, les attaques répétées qui atteignent la dignité humaine ne sont pas chose nouvelle. le jeune Charles Bovary, par son accoutrement de paysan normand et sa balourdise, avait subi la risée de sa classe. En 1857, Gustave Flaubert décrit ce harcèlement scolaire dans le premier chapitre de son roman pour brosser les faiblesses de caractère du futur mari d'Emma. L'expansion de l'usage des outils numériques, jusque dans les mains d'enfants de plus en plus jeunes, a incontestablement donné à ce harcèlement scolaire, que vous qualifiez de cyberharcèlement, une ampleur et conduit à des modes opératoires nouveaux et toujours plus pernicieux, qui exigeaient que le Sénat s'en préoccupât.

Les premiers travaux parlementaires sur ce sujet ont été entrepris il y a une dizaine d'années, mais le rapport qui sert de prétexte à ce débat dresse un bilan nouveau, utile et alarmant de l'étendue du phénomène, et prévoit le cadre d'une politique nationale qui mérite d'être discuté dans cet dans cet hémicycle. Nous partageons l'idée que les établissements d'enseignement et les équipes éducatives, dans leur intégralité, doivent être au coeur de la lutte contre ce harcèlement, même si ce dernier peut se poursuivre à la maison à cause de la domination toujours plus despotique des réseaux dits « sociaux De nouvelles compétences pourraient certainement être acquises par ces équipes ; des formations nouvelles devront sans doute leur être proposées. Néanmoins, encore une fois, ces récentes exigences nous imposent de réfléchir collectivement à la place de l'école dans la société et à la mission donnée à l'enseignant. La mission de l'école n'a jamais été de transmettre uniquement des savoirs et des connaissances. Celle-ci a toujours contribué à l'émancipation individuelle, à la diffusion d'une morale républicaine. En un mot, elle se devait d'éduquer, dans le sens latin du verbe, c'est-à-dire de former des esprits. Alors que les cadres moraux de nos sociétés vacillent, la tentation est grande de demander à l'école d'apporter, par l'éducation, des remèdes à tous les maux qui nous accablent. Souvent, y compris dans cet hémicycle, nous y cédons en ajoutant des lignes aux programmes des élèves et de formation des professeurs. Cette pratique risque fort de transformer le code de l'éducation en un cahier de doléances. En l'occurrence, il n'est pas absurde de confier à l'école une mission particulière en matière de cyberharcèlement scolaire, mais il ne faudrait pas qu'elle s'ajoute à toutes celles qui incombent depuis peu aux enseignements. Le rapport dont nous débattons recommande avec raison la reconstitution, dans les établissements, d'équipes pluridisciplinaires composées de médecins, de psychologues et d'assistantes sociales, pour assurer cet indispensable travail d'accompagnement. La deuxième préconisation forte de ce rapport, dont nous partageons totalement l'esprit, concerne les réseaux dits « sociaux ». Nous discutons de ce rapport, alors que les révélations de Frances Haugen, ancienne ingénieure de Facebook chargée de « l'intégrité civique »- ! -, jettent une lumière crue crue sur ce qui constitue la banqueroute morale de ce réseau de destruction sociale. Les machines algorithmiques qui sont au coeur de ces réseaux sont paramétrées pour retenir l'attention. Or cette captation est l'objet même de leur modèle économique. Les réseaux qui les utilisent n'ont donc aucun intérêt à les réguler : ils sont complices de leur propagation. Le psychiatre Serge Tisseron considère que ces réseaux sont des produits toxiques, et qu'il faudrait les réglementer comme des aliments dangereux pour la santé. Au lieu de cela, nous nous contentons de les appeler à la raison et nous leur demandons, par faiblesse, d'organiser eux-mêmes leur régulation. Ainsi, la loi du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information, qui confie au Conseil supérieur de l'audiovisuel la mission d'analyser le fonctionnement des algorithmes des plateformes n'est pas appliquée, faute d'un régime de sanctions contraignant. Le Sénat l'a déjà affirmé à plusieurs reprises, et je le redis avec force devant vous : puisque nous convenons tous qu'il est urgent d'agir sur les vecteurs du cyberharcèlement, aucune évolution positive n'est à attendre de ces entreprises tant que nous ne nous attaquerons pas à leur modèle économique. Nous devons le faire urgemment pour la santé psychique et morale de nos enfants. La parole

Il est urgent que chacun d'entre nous prenne conscience de cette réalité et mesure le drame individuel et collectif que le harcèlement représente aujourd'hui pour notre école.

Sur la plateforme TikTok, le hashtag #Anti2010 a prospéré, et des vidéos invitent les jeunes à s'en prendre à ces élèves de En 2020, à la suite du confinement et de la fermeture des établissements scolaires, le cyberharcèlement s'est dramatiquement accru. La plateforme d'écoute de l'association e-Enfance a ainsi enregistré une hausse de 30 % des appels, ce qui a entraîné deux fois plus de signalements. Aucun établissement, aucune région, aucune catégorie sociale ne sont épargnés. Face à cette réalité, le corps enseignant s'estime souvent désarmé. Sont en cause le manque de formation et la difficulté à identifier les cas. C'est pourquoi il me paraît primordial d'intégrer dans la formation initiale et continue des enseignants une sensibilisation à l'empathie et à la détection des situations de harcèlement. Je rappelle que les conséquences du harcèlement sont graves. Celui-ci accroît le risque d'entrer dans la délinquance criminelle, d'adopter des conduites à risques et peut pousser la victime au suicide. Mardi, dans les colonnes de était évoqué le cas de Chanel, 12 ans, victime de harcèlement ayant mis fin à ses jours le 30 septembre dernier.

avancées. De nombreuses actions ont été engagées par le ministère de l'éducation nationale : la publication de guides à l'attention des équipes éducatives, l'instauration d'une ligne d'écoute téléphonique nationale, la création d'un site internet proposant des ressources aux enseignants et aux parents, la liste n'étant pas exhaustive autant de dispositifs qui visent à protéger l'intérêt supérieur de l'enfant et de l'adolescent dans la construction de son identité et dans sa formation scolaire. Tous les ministres de l'éducation nationale ont poursuivi cette politique publique. Des partenariats entre les services de police et de gendarmerie, les équipes enseignantes et le personnel médico-social existent. Les départements et les régions mènent également très souvent des campagnes de sensibilisation et de formation de leurs agents. les associations de victimes, elles aussi, oeuvrent chaque jour auprès des victimes- je souhaite saluer ici la mobilisation de tous les acteurs. Malgré tous ces efforts et tous les instruments qui sont déployés, la lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement se révèle aujourd'hui imparfaite sur plusieurs points. D'abord, si les outils à la disposition des pouvoirs publics sont nombreux, ils sont peu connus. Ensuite, l'arsenal juridique existant est souvent inadapté face au cyberharcèlement. Les enseignants sont par ailleurs trop peu formés pour faire face à ces situations. Faute d'une formation adaptée, seuls 35 % d'entre eux se sentent armés pour gérer une situation de harcèlement. 83 % des enseignants indiquent n'avoir jamais reçu de formation consacrée à la prévention et à la gestion du harcèlement. Ils sont tout aussi nombreux à estimer que cette lutte doit être considérée comme un enjeu de santé publique. un dernier point, le manque de moyens humains et financiers dans les établissements. La lutte contre le harcèlement implique des moyens humains mobilisant l'ensemble de la communauté éducative. L'intervention de tiers extérieurs à l'établissement figure parmi les initiatives intéressantes mises en oeuvre, mais cette intervention a un coût difficile à assumer, notamment pour les collèges.

prévenir, détecter, traiter. Afin de mieux prévenir les cas de harcèlement, nous recommandons notamment de faire un point systématique, à chaque rentrée, dans chaque académie, sur la qualité du climat scolaire de manière systématique, au niveau de l'académie les faits de harcèlement et en présenter les suites devant le conseil d'administration de l'établissement. Pour détecter les cas de harcèlement, il faut intégrer dans intégrer dans la formation des enseignants une sensibilisation à l'empathie et à la détection des situations de harcèlement ; mesurer précisément par cycle scolaire et par région l'ampleur du harcèlement scolaire. Pour traiter rapidement et efficacement les cas qui se présentent, il faut continuer à développer les travaux d'intérêt général et les stages de citoyenneté traitant de harcèlement pour les enfants harceleurs

Le dixième et dernier principe de la Déclaration universelle des droits de l'enfant nous rappelle que l'enfant doit être protégé contre toute forme de discrimination. C'est dans cet unique but qu'il nous incombe de lutter sans relâche contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement, qui remettent en cause le droit essentiel de l'enfant à s'instruire

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le cyberharcèlement s'est de nouveau invité dans le débat public avec le hashtag #Anti2010. Alors que nous sommes concentrés sur la gestion de la crise sanitaire depuis de longs mois maintenant, ce déferlement de haine en ligne- j'utilise ce mot volontairement -est venu mettre encore plus en évidence le mal-être des jeunes, qui s'est accru depuis le début de la pandémie. Si la France demeure dans la moyenne des pays européens concernant le harcèlement et le cyberharcèlement, les politiques publiques mises en place sont extrêmement récentes : elles n'ont qu'une dizaine d'années, alors que dans d'autres pays le problème est pris à bras-le-corps depuis des décennies.

ont d'ailleurs, sur ce sujet, un grand rôle à jouer, rôle d'autant plus important que le harcèlement se met en place, aussi, sur les réseaux sociaux, qui n'offrent plus aucune période de repos aux jeunes victimes. Les problèmes de l'école se retrouvent le soir sur les réseaux, et vice versa. Les statistiques varient, selon ce que l'on intègre dans la notion de harcèlement. Si je me réfère à l'excellent et très complet rapport de notre collègue Colette Mélot pour la mission d'information à laquelle j'ai participé, au moins 6 % des élèves subiraient une forme de harcèlement scolaire, soit plus de 800 000 jeunes chaque année. Ce chiffre colossal est inquiétant quand on sait que le harcèlement peut conduire à des troubles du comportement, plus ou moins graves, des dépressions, jusqu'à des gestes suicidaires dont certains aboutissent. Je pense, par exemple, à ce jeune marseillais de 13 ans, atteint de troubles « dys », qui a fait deux tentatives de suicide à la suite au harcèlement qu'il a subi,

potentiels pour espérer résoudre le problème. Ce sont toutes les valeurs qui traversent non seulement l'école, mais aussi la famille et la société tout entière qui doivent être questionnées. Selon Catherine Blaya, une professeure qui dirige des travaux de recherche sur le sujet, les pays les plus concernés par la violence sur les réseaux sociaux sont aussi ceux où il y a le plus de violence dans la société. Le Le fond du problème me semble être là. Je note d'ailleurs avec satisfaction que les préconisations du rapport en matière de prévention sont les plus nombreuses. Dans beaucoup de domaines, mieux vaut prévenir

En travaillant sur l'empathie et la réflexion des élèves harceleurs et de leurs familles, les modèles suédois et norvégien, appliqués dans de nombreux autres pays, ont fait leurs preuves. Ils sont plus favorables à la création d'un sentiment de communauté entre les élèves, et entre les élèves et l'équipe éducative.

c'est vrai, un cadre strict et des sanctions si nécessaire. Pour cela, le personnel encadrant doit être formé et engagé sur cette cause. C'est un préalable indispensable sur lequel notre pays doit, me semble-t-il, encore travailler, y compris sur les temps périscolaires où les collectivités ont un rôle à jouer. Le décloisonnement est plus que jamais

Elles peuvent se décliner en mesures concrètes, telles que des travaux de groupe ou des jeux de rôle, pour inciter témoins et victimes à manifester leur réprobation, résoudre les éventuels conflits et se mettre à la place des victimes. l'empathie. On sait que le cyberharcèlement est plus fréquent chez les écoliers du primaire, avec 14 % de victimes parmi les élèves du CE2 au CM2. Peut-être faudrait-il mieux prévenir les familles et limiter davantage le recours à internet à ces âges.

J'étais hier à Frévent, petite commune du Pas-de-Calais, pour participer à la marche blanche organisée en la mémoire de Chanel, une enfant de 12 ans qui a mis fin à ses jours parce qu'elle était harcelée, violemment et depuis trop longtemps. Permettez-moi d'associer l'ensemble de notre assemblée au soutien que j'exprime à l'endroit de sa famille et de ses proches. Avec notre rapporteure, Colette Mélot, dont je tiens à saluer la très forte implication, ainsi d'ailleurs que celle de tous les membres de la mission, me semble-t-il, utilement oeuvré en faveur d'une détection plus précoce du harcèlement, d'un suivi mieux assuré et d'un traitement plus efficace, avec la volonté de mettre un terme à ce fléau.

Elles sont classées par grande priorité et par ordre chronologique, avec l'indication systématique de l'entité qui en a la responsabilité, du vecteur juridique à mobiliser et du calendrier de mise en oeuvre.

Chacun voit bien à quel point le harcèlement scolaire représente pour notre société un drame, individuel et collectif, qu'il est plus que jamais urgent de combattre, tant il sape insidieusement les fondements de notre bien vivre ensemble. Le mouvement de harcèlement à l'encontre des élèves de sixième nés en 2010, survenu à la mi-septembre dans nos collèges, en montre encore, s'il en était besoin, la malheureuse actualité, tout autant que le caractère proprement irrationnel. Si la mobilisation est réelle et si les outils de sensibilisation existent, le dispositif actuel contre le harcèlement scolaire pèche encore dans le suivi, qui n'est pas suffisamment assuré. Mon intervention portera donc tant sur le fond que sur la forme de cette mise en oeuvre. Sur le fond, et sans revenir sur les points que mes collègues ont déjà pu aborder, j'ai principalement deux séries de questions à évoquer devant vous. La première série porte sur les moyens nécessaires pour lutter contre le harcèlement et leur renforcement indispensable. Nos auditions l'ont amplement montré : tant la prévention que la détection suppose que les moyens humains de l'éducation nationale soient à la hauteur. Nos déplacements sur le terrain dans deux collèges, à Melun et à Douvrin, ont permis de constater la forte implication des personnels, tout autant que l'efficacité de leur action au quotidien. Cette action est menée en lien étroit avec les autres partenaires publics que sont la police, la gendarmerie et la justice, ainsi qu'avec les associations. Le succès en la matière du collège de Melun, en particulier, semble autant dû à l'implication dévouée de ses personnels qu'aux moyens supplémentaires dont il bénéficie en tant que collège Les professeurs, dont les heures de cours sont pondérées, utilisent celles qui leur restent pour organiser des temps d'équipe, permettant d'échanger et, donc, d'identifier beaucoup plus rapidement les situations anormales, tout en maintenant un climat scolaire serein. La mobilisation générale contre le harcèlement scolaire suppose donc bien que la gestion de ces moyens humains se fasse de façon plus fine qu'actuellement. Il faut éviter un turn-over trop rapide afin que les personnels en place disposent du temps nécessaire pour asseoir leur légitimité et leur positionnement au sein de l'équipe éducative. Les premières indications concernant le projet de budget pour 2022 paraissent montrer des créations de postes d'infirmiers scolaires, d'assistants sociaux et de CPE dans l'enseignement secondaire, avec notamment l'ouverture de 300 postes de CPE et de 50 postes d'assistants sociaux et infirmiers. Si ces ouvertures de postes répondent en partie à notre attente de plus de moyens et de personnels dans les établissements, encore faut-il que les postes ainsi ouverts soient effectivement pourvus ... Pour cela, madame la secrétaire d'État, il faudra veiller à leur attractivité. Par ailleurs, Par ailleurs, s'agissant des assistants sociaux et des infirmiers, les besoins actuels sont importants, surtout au regard du faible nombre de postes ouverts. Ainsi, les 50 postes d'assistants sociaux ou d'infirmiers prévus au budget ne représentent qu'un petit « demi-poste » par département absolument insuffisant, eu égard aux attentes de la communauté éducative et des parents. Madame la secrétaire d'État, au titre du suivi vigilant qui sera le nôtre, et que notre rapporteure a rappelé, nous attendons des éclaircissements sur cette question cruciale de l'accroissement, indispensable et significatif, des moyens de lutte contre le harcèlement scolaire.

Vous le savez, une partie de la lutte contre le cyberharcèlement véhiculé par les réseaux sociaux passe par une action déterminée au niveau communautaire, qui viserait à leur imposer des ou diffuser la pratique du, comme l'a rappelé notre rapporteure. Lors de nos auditions, nous avons bien constaté que les représentants de ces réseaux ne réagissaient réellement que sous contrainte, quand ils étaient soumis à une forte pression tant politique que médiatique. À ce sujet, je continue de regretter que l'un de ces réseaux, et pas des moindres puisqu'il s'agit de Twitter, n'ait pas pu ou pas voulu participer à notre table ronde du 23 juin dernier. Madame la secrétaire d'État, votre collègue secrétaire d'État aux affaires européennes a indiqué voilà une semaine, lors d'une audition à l'Assemblée nationale, que le programme détaillé de cette présidence serait dévoilé par l'exécutif le 1 décembre prochain. Pouvez-vous nous rassurer dès à présent, et clairement, quant à la suite positive que vous allez réserver à cette demande pressante ? Ces priorités figureront-elles bien dans la feuille de route du prochain semestre européen dont vous aurez la charge ? Enfin, et pour conclure mon propos, je sais que vous avez lu le rapport de notre mission d'information. Nous l'avons voulu opérationnel. Les choses sont dites, les recommandations séquencées dans le temps, les vecteurs juridiques précisés, ainsi que les acteurs publics ou privés en charge de leur mise en oeuvre. L'école ne doit pas être un lieu de souffrance. Elle forme notre jeunesse pour en faire les adultes-citoyens de demain, et je vous sais attachée à ces valeurs. Alors, comme mes vingt-deux collègues membres de la mission d'information, nous espérons que, avec le ministre Jean-Michel Blanquer, vous agirez vite et bien. Saisissez-vous de ce rapport ! La mission a bien travaillé, tout y est ! C'est une question de volonté politique.

à remercier Mme Colette Mélot, rapporteure de la mission d'information, et Mme Sabine Van Heghe, sa présidente, pour la conduite des travaux et l'écriture des conclusions qui viennent d'être publiées sur ce sujet essentiel.

Tous les ans, plus de 700 000 enfants sont cassés, abîmés par le harcèlement scolaire. Ils se débattent au milieu de leurs cauchemars, de leurs peurs, de leur confiance en eux, en l'autre qui à chaque fois s'envole un peu plus. » Tel est le constat, effrayant, que dresse l'association Les Papillons sur son site internet. Cette structure, présente dans plusieurs départements, dont le Finistère, vise à libérer la parole des enfants victimes de maltraitances. Elle est d'ailleurs citée, comme d'autres structures impliquées dans ce domaine, dans le rapport de la mission. L'« affaire Mila » a aussi récemment marqué les esprits. L'histoire de cette jeune fille, victime d'un raid numérique, sujette à des menaces de mort, des appels au viol, des insultes, a remis en lumière les effets dramatiques du harcèlement, en l'occurrence du cyberharcèlement, et ses conséquences bien réelles. En juillet, onze prévenus ont été condamnés. Le Le harcèlement est bien un fléau, qui se retrouve à tout âge et dans tous les champs de la vie sociale : à l'école- cour de récréation, classe ou vestiaire -, au travail, dans la sphère familiale et dans les espaces publics, en ligne ou dans la rue.

avec des conséquences sur le long terme, entraînant des traumatismes profonds et des fragilités durables. Aussi de nombreuses actions sont-elles menées. La loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance consacre, en son article 5, le droit à une scolarité sans harcèlement, reconnaissant ainsi la gravité de cette forme de violence scolaire. scolaire. L'encadrement de l'utilisation des portables dans les établissements scolaires vise ce même objectif. Un numéro contre le harcèlement scolaire est disponible, de même que contre le cyberharcèlement. Des ressources pédagogiques ont été élaborées. Plusieurs « élèves ambassadeurs », en collège et en lycée, peuvent être nommés. Des référents ont été mis en place. Le travail avec les associations se poursuit et se renforce. Mais le phénomène a pu connaître un rebond durant la période de confinement, comme l'a rappelé le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports voilà quelques mois. Il est aussi absolument nécessaire d'intervenir à trois niveaux. En amont, par une éducation aux médias renforcée tout au long de la scolarité et une prévention dans le milieu scolaire, notamment par la sensibilisation des plus jeunes aux conséquences du cyberharcèlement et une information sur les accompagnements existants. Par une prise en charge rapide des victimes de harcèlement ou cyberharcèlement dès les premiers « signaux faibles », ce qui implique de savoir détecter ces derniers rapidement, avec le partage de dispositifs simples, d'outils identifiés par les enfants, par les familles et par toutes les équipes éducatives. Il est indispensable que des personnes ressources, de proximité et de confiance, soient connues des enfants pour plus de réactivité dans l'accompagnement. En aval, enfin, par un accompagnement des harceleurs et un renforcement de l'efficacité de la réponse pénale à l'égard des auteurs. La sanction doit, de toutes les façons, s'accompagner d'une prise de conscience de l'agresseur. Les plateformes ont évidemment un rôle de coopération primordial à jouer, en lien avec les pouvoirs publics. Leur responsabilité est engagée. Les signalements doivent pouvoir se faire rapidement, puis être traités avec la même célérité. Il s'agit bien entendu d'un sujet global puisque, si le cyberharcèlement franchit les murs des établissements, les politiques de régulation appellent aussi à dépasser les frontières étatiques. En fin d'année dernière, l'Unesco et le ministère français de l'éducation nationale avaient organisé une conférence internationale sur la lutte contre le harcèlement Cette problématique pourra être abordée lors de la présidence française de l'Union européenne. Le Gouvernement a récemment annoncé la généralisation sur tout le territoire du programme de lutte contre le harcèlement à l'école Phare, sur la base de l'expérimentation menée, depuis deux ans, dans six académies. En cette rentrée, un projet de loi visant à mieux protéger les victimes, en soignant aussi les harceleurs, va être discuté au Danemark. Cette approche était préconisée par la méthode de la « préoccupation partagée », développée dès le début des années 1980 en Suède par Anatol Pikas ; elle est aujourd'hui utilisée avec succès en Finlande, en Australie et au Canada. De la même manière, pour lutter contre le harcèlement scolaire, les Finlandais ont inventé une méthode appelée KiVa. Échangeons donc sur nos dispositifs de lutte afin de combattre, ensemble, ce fléau

traduisait l'idéal républicain : l'éducation remplit une mission fondamentale. À ceux qui affirmaient que les criminels étaient responsables de leur état, il répondait depuis ces travées : « Tout homme coupable est une éducation manquée qu'il faut refaire. L'école dispense le premier remède contre la violence, par l'apprentissage du civisme et de la citoyenneté. À côté des règles de grammaire et de conjugaison, des jalons de l'histoire de France et de l'algèbre, l'acquisition de compétences psychosociales est indispensable à la cohésion d'une communauté, à l'échelle d'une école, comme à l'échelle comme à l'échelle d'une nation. À l'origine de tout harcèlement se trouve bien souvent une défaillance d'empathie de la part d'individus incapables de se mettre à la place des autres, de se représenter les conséquences de leurs actes, nourris par un sentiment de toute-puissance. Du côté des victimes, la peur, la honte et, souvent, une fausse culpabilité paralysent la parole. Les harceleurs s'attaquent en général à des élèves pacifiques, isolés, plutôt introvertis, instaurant un rapport de force inégal et un mécanisme odieux de violence. L'étendue du phénomène, sa banalisation insupportable et l'augmentation des cas de cyberharcèlement font de ce fléau un fait de société, qu'il faut que nous combattions de toute urgence. C'est précisément l'objectif que s'est donné le groupe Les Indépendants - République et Territoires,

Comme l'explique le rapport présenté le 23 septembre dernier, le harcèlement scolaire engendre des conséquences dramatiques pour les victimes, à commencer par le désengagement scolaire selon les enquêtes nationales de 2010 et 2011, le harcèlement est à l'origine de 25 % des cas d'absentéisme chronique. Il est responsable d'une très forte augmentation des risques de dépression et de suicide. L'état de stress permanent dans lequel il plonge l'élève n'épargne aucune sphère de sa vie, à court terme, mais aussi à très long terme. Malheureusement, dix ans d'actions des gouvernements successifs n'ont pas permis d'éradiquer le problème. De nombreux outils existent, et c'est pourquoi la mission d'information s'est intéressée à l'application sur le terrain des dispositifs déployés.

Cela passe par une mobilisation générale de la communauté éducative, appuyée par les parents d'élèves et les associations. Nous devons aussi placer les responsables des réseaux sociaux face à leur responsabilité.

de harcèlement une stratégie de sortie de crise lui permettant de reprendre le contrôle de la situation et de briser la spirale du harcèlement, renforçant dans un même temps sa confiance en

Madame la secrétaire d'État, j'aimerais que vous considériez cette proposition de former le personnel compétent en matière de lutte contre le harcèlement scolaire aux méthodes visant à renforcer l'affirmation de soi chez les élèves qui en sont victimes. La parole est à Mme Sabine

tout comme les précédents orateurs, je voudrais moi aussi saluer le travail accompli par la mission d'information, sa présidente et sa rapporteure. En tant que membre de cette mission, je peux témoigner du fait que personne n'est ressorti indemne des auditions auxquelles nous avons pu prendre part. Le harcèlement scolaire débute dès l'école élémentaire, parfois même dès la maternelle. Or l'enjeu n'est pas seulement d'y faire face par la voie des sanctions et de la judiciarisation. s'agit aussi de se donner, ou plutôt de se redonner les moyens de mener un travail au sein de l'école afin d'y réinstaurer un climat susceptible de permettre à chaque enfant de se sentir suffisamment en sécurité pour s'investir dans les activités et les contenus scolaires qui lui sont proposés.

de directeurs d'école formés à ces problématiques, il intervient lorsque les équipes, dans les classes, ne sont plus en mesure de gérer une situation en interne. membres de ce groupe prennent en charge l'élève harcelé, ainsi que son ou ses harceleurs, pour les aider à trouver, avec eux, les ressources pour changer les choses, pour les responsabiliser, les rendre acteurs et les inciter à trouver des solutions qui permettront d'éviter le recours à la sanction. Cette méthode vise à « redonner une place centrale au respect, à l'empathie, une chance à la fois à l'agresseur et à l'agressé », à « sortir de la spirale infernale " violences-sanctions-violences comme l'explique Fabienne Schlund, inspectrice de la circonscription qui a pris l'initiative de créer ce groupe, à la suite de son travail de recherche et de sa thèse. Les actions mises en oeuvre dans les classes par son équipe ont permis de juguler ces phénomènes dans les écoles primaires de son secteur. Mais pour mener ces actions de prévention et de remédiation,

comme les aider à faire face aux difficultés qu'ils rencontrent dans la gestion de leurs classes et celles, surtout, de leurs élèves dépassés par les attentes de l'école ou pris dans la spirale du harcèlement en tant que victimes ou auteurs.

disposaient de moyens humains qui leur permettaient d'assurer une présence régulière dans les écoles, notamment rurales, et de mettre en oeuvre des actions de prévention et de remédiation auprès des élèves, d'accompagner et de soutenir leurs parents et leurs enseignants. Aujourd'hui ces structures ne sont plus en mesure, par manque de postes et de personnels, de remplir leurs missions. Les enseignants, notamment ceux qui enseignent dans des territoires éloignés de structures médico-psycho-pédagogiques ou socio-éducatives, n'ont ni la formation ni la disponibilité nécessaire pour faire face, seuls, à ces phénomènes qui explosent partout, en n'épargnant aucun territoire ni aucune classe sociale.

le rapport de notre mission d'information a un mérite, celui d'attirer vivement l'attention sur un phénomène de plus en plus répandu, multiple dans ses modalités et ses conséquences dramatiques. Depuis le 1 janvier 2021, Nous sommes tous partisans d'une mobilisation générale. Les recommandations du rapport, pragmatiques, ne peuvent qu'être approuvées et il est bon qu'un échéancier accompagne ces préconisations très concrètes. Il est inutile de revenir sur les constats d'un fléau dont la violence s'est accentuée avec celle des réseaux sociaux. inutile de revenir sur l'insuffisance de l'action actuellement déployée : l'abaissement continu de l'âge de possession du premier smartphone en démontre toutes les limites. Les élèves de l'école primaire sont de plus en plus largement concernés, aux âges charnières du début de la construction de l'identité. Ce danger qui menace nos enfants ne peut être ni analysé ni combattu sans une prise en compte globale de l'environnement dans lequel il se situe, sans la volonté de ne pas s'y plier passivement, par fatalisme, impuissance ou absence de volonté politique. Toutes les actions proposées doivent s'inscrire dans une telle perspective politique générale. Des effets d'annonce sans lendemain, de la part de l'exécutif, ne seraient pas à la hauteur des défis qui sont devant nous. Il faut commencer par la prise de conscience en s'adressant aux Français de manière simple, claire et directe. J'espère que le débat d'aujourd'hui y contribuera. Le cyberharcèlement est une thématique à l'intérieur de la problématique numérique. Il sera difficile de renforcer durablement les défenses de nos enfants si nous n'acceptons pas de voir que le système numérique tout entier est organisé pour les rendre réceptifs l'ensemble des moyens utilisés par les réseaux relèvent de l'addiction et des circuits de la récompense. Ils doivent être traités comme tels dans notre pays et de nouveaux chantiers s'ouvriront Les moyens de contraindre les réseaux sociaux à plus de vigilance existent. Le rapport souligne que la présidence française de l'Union européenne est une occasion à ne pas rater. Toutefois, je ne suis pas persuadé que les grandes plateformes redoutent particulièrement cette échéance. L'Europe n'est pas toujours unanime sur ces sujets et elle se révèle trop souvent frileuse. Les combats seront compliqués et ardus, du fait, notamment, de la réactivité des grandes plateformes. Renforcer leurs obligations exigera un volontarisme national, européen et mondial sans faille. Pour ce qui concerne la responsabilité parentale, il faut se garder des culpabilisations excessives. Il faut prendre conscience, là encore, que le rapport des parents aux réseaux sociaux est significatif pour leurs enfants. Pour les parents, la question est simple : qui acceptent-ils de voir entrer dans leur foyer ?

il faut aller au-delà d'une simple sensibilisation « soft ». Je suis favorable à ce que des images de publicité fortes, voire choquantes, rendent le message d'alerte officiellement plus présent à nos concitoyens. L'exemple peut venir de certains pays voisins. Il est impératif de compléter ainsi les outils actuels, trop dispersés, trop bureaucratiques, en tout cas inconnus du grand public. Ce débat est aussi un appel à une citoyenneté et un civisme exigeants, aux plans individuel et collectif. C'est d'une vision républicaine, où la raison et les lumières l'emportent, que nous avons besoin, pas d'un usage obscurantiste où la violence sous toutes ses formes s'associe au complotisme dans un anonymat délétère. matière pénale, les sanctions restent très largement insuffisantes. L'effet de groupe, la puissance du collectif conduisent à négliger la responsabilité de ceux qui se taisent et n'osent s'opposer ; et cette insuffisance accentue encore la violence de la relation entre harceleur et harcelé. Les peines, facteurs d'exemplarité, ne sauraient épargner les participants qui, de manière abusive, s'estiment passifs. Notre lutte contre le harcèlement scolaire ne peut qu'être consensuelle, en dépassant les préjugés idéologiques et les excuses sociologiques.

parce qu'elles ont des responsabilités éducatives, les collectivités territoriales peuvent jouer un rôle accru dans la proximité et la prévention. Le Sénat, chambre des territoires, y sera attentif !

Le harcèlement et le cyberharcèlement sont des sujets prioritaires. Ils concentrent l'attention du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Jean-Michel Blanquer,

La cyberviolence ne peut plus être déconnectée des violences subies dans le cadre scolaire, puisqu'elle se propage très souvent par la diffusion entre pairs. Nous le savons : combiné aux réseaux sociaux et aux outils de communication de jeux

#Anti2010, qui a émergé progressivement sur des plateformes de jeux en ligne avant de contaminer certains réseaux sociaux, et qui nous a conduits à intervenir rapidement en lançant un autre hashtag : #BienvenueAux2010.

Depuis quatre ans, notre ministère a placé la lutte contre le harcèlement scolaire en tête de ses priorités, en conduisant une politique publique volontariste et ambitieuse de lutte contre toutes les formes de harcèlement.

car les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Je le disais précédemment : le harcèlement, aujourd'hui, c'est aussi le cyberharcèlement.

par tous, le phénomène serait déjà en partie jugulé. Notre responsabilité, c'est aussi de sensibiliser et d'accompagner. C'est la raison pour laquelle nous développons une approche partenariale avec les différents réseaux sociaux afin d'anticiper et d'endiguer les phénomènes viraux.

et leurs initiatives doivent être valorisées. Le traumatisme des victimes est réel et sa réduction devient un enjeu de santé publique. la puissance publique ne peut pas tout et les associations de terrain font un travail remarquable dans ce domaine : elles sont à même de nous aider. Aujourd'hui, plus d'un élève de sixième sur deux dispose d'un compte sur un réseau social. Il est donc nécessaire d'apprendre aux enfants à communiquer sur ces plateformes. C'est aussi la mission de l'éducation aux médias et à l'information, dès la fin de l'école primaire. En effet, nos enfants doivent absolument avoir les clefs pour naviguer dans cet univers : la prise de conscience et le travail des élèves par eux-mêmes sont des éléments décisifs pour combattre durablement le harcèlement. Je tiens également à témoigner personnellement de l'amélioration des pratiques sur le terrain, pour le repérage et le traitement des situations de harcèlement et de cyberharcèlement dans les écoles, les collèges et les lycées.

La sensibilisation et la formation des acteurs de l'école pour écouter, répondre, alerter et réparer doivent permettre aux enfants et aux adolescents de se sentir de nouveau en confiance. Il n'est pas question de s'arrêter là, car beaucoup reste à faire. Chaque situation de harcèlement est une situation de trop ; mais, avec les familles, nous devons trouver les voies de l'apaisement sur ces sujets et permettre à chaque élève victime d'évoluer sereinement avec ses camarades, dans la sphère scolaire comme dans la sphère privée. C'est un enjeu de protection de l'intégrité morale et physique de nos élèves, face à un phénomène qui, je le disais en préambule, peut avoir des répercussions terribles